Les discussions ont été dominées par la question de la lutte contre le changement climatique. Comme ils en étaient convenus au mois de juin dernier, les chefs d'État et de gouvernement ont endossé l'objectif de la neutralité carbone d'ici à 2050.

puis un peu plus d'une vingtaine à l'été, a obtenu que l'unanimité se fasse autour de cet objectif. En s'engageant à devenir le premier continent neutre en carbone en 2050, l'Union européenne donne un signal clair sur son ambition.

sein de son mix énergétique et du coût élevé de la transition pour la Pologne. Cette exemption temporaire n'a pas conduit à repousser l'adoption de l'objectif collectif

Un certain nombre de propositions ont été faites en ce sens par la Commission dans son Pacte vert. J'insisterai sur le mécanisme d'inclusion carbone aux frontières, essentiel

une clarification utile. J'y reviendrai si vous le souhaitez. Enfin, le Conseil européen a invité la Commission à préparer en temps utile, avant la COP26 de Glasgow, au terme d'une analyse d'impact approfondie, la proposition relative à la mise à jour de la contribution déterminée au niveau national (CDN)

un seul élément du triangle organisationnel européen. Alors que les institutions se préparent à l'organisation de cette conférence- nous attendons une communication de la Commission 2020, ainsi qu'une résolution du Parlement européen -, le Conseil européen a demandé à la future présidence croate d'établir une position du Conseil sur le contenu, la portée, la composition et le fonctionnement d'une telle conférence.

en particulier nous assurer que l'augmentation de la PAC repose non seulement sur le second pilier, comme c'est le cas aujourd'hui, mais également sur le premier. Je le redis devant vous

l'approfondissement de l'Union économique et monétaire, la poursuite des travaux sur le mécanisme européen de stabilité, le renforcement de l'union bancaire et le budget de la zone euro. Le Président de la République a Le Président de la République a souligné que si les progrès sur ces différents sujets étaient certains, ils restent largement insuffisants, en particulier parce que nous voudrions que ces outils, au service notamment de la zone euro, soient non seulement des instruments de convergence, mais aussi de stabilisation. nous avons terminé cette longue réunion par une session en format « article 50 », puisque nous étions au lendemain des élections britanniques. La nette victoire de de Boris Johnson nous permet d'entrevoir une sortie ordonnée du Royaume-Uni après plus de trois ans de débats complexes. Nous avons surtout, pendant cette réunion, posé les principes qui guideront la négociation de la relation future

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, au moment même où se tenait le Conseil européen des 12 et 13 décembre, le Royaume-Uni nous adressait enfin un message clair sur le Brexit. Avec cette victoire sans appel de Boris Johnson, le peuple britannique nous dit enfin ce qu'il veut, après plus de trois ans d'une incertitude qui a affaibli l'Europe dans son ensemble. Nous regrettons le Brexit, contresens historique majeur, mais nous respectons le choix du peuple britannique. De nouvelles négociations sur la relation future vont s'ouvrir. Des questions épineuses se poseront. Le compromis trouvé sur la frontière irlandaise, le fameux « », sera tout sauf simple à mettre en oeuvre. Je le dis avec force : l'intégrité du marché unique européen doit être préservée. Le groupe de suivi sur le Brexit, coprésidé par les présidents Cambon et Bizet, a révélé les risques pesant sur l'intégrité territoriale du Royaume-Uni du fait du Brexit.

La question irlandaise elle-même pourrait rebondir, alors que les unionistes font partie des grands perdants de cette élection. Notre groupe de suivi a enfin pointé le risque d'un dumping fiscal, social et réglementaire aux frontières de l'Europe, avec le fameux « Singapour sur sur Tamise ». La forte légitimité dont bénéficie désormais Boris Johnson pourrait l'inciter à frapper vite et fort. Restons vigilants dans la nouvelle phase de négociation. La relation future devra maintenir les intérêts européens et aboutir à un degré élevé de coopération avec le Royaume-Uni, en particulier sur les plans de la sécurité et de la défense. J'invite le Gouvernement à profiter de la célébration des dix ans du traité de Lancaster House, en novembre prochain, pour obtenir des avancées fortes en la matière. La commission des affaires étrangères va préparer cette échéance avec son homologue britannique. La défense européenne, justement, doit être une priorité. Le budget du Fonds européen de la défense (Fedef) est « une ligne rouge pour la France », nous avez-vous dit ici même, madame La commission des affaires étrangères et de la défense estime que nous ne pouvons pas manquer le tournant du Fedef. Le Conseil européen a rappelé son opposition aux activités de forage illégales de la Turquie dans la zone économique exclusive de Chypre et a estimé que le protocole d'accord entre la Turquie et la Libye sur la délimitation en mer Méditerranée violait le droit. Je tenais à réaffirmer ici sans équivoque notre solidarité avec la Grèce et Chypre en ce qui concerne ces actions de la Turquie. Madame la secrétaire d'État, l'Union a une nouvelle page de son histoire à écrire. Nous comptons sur vous pour qu'elle soit ambitieuse. Très bien

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le dernier Conseil européen de l'année s'est tenu dans un paysage institutionnel renouvelé, marqué par l'entrée en fonction de la nouvelle Commission européenne et de celle de Charles Michel à la tête du Conseil européen. Si la présentation par la Commission de son Pacte vert a occupé une part significative des échanges, d'autres sujets qui intéressent plus particulièrement la commission des finances ont été abordés. Tout d'abord, ce Conseil européen était une échéance très attendue en vue des négociations du prochain cadre financier pluriannuel (CFP) pour les années 2021 à 2027. Or force est de constater que la dernière proposition de la présidence finlandaise, établissant le budget européen à 1,07 % du revenu national brut (RNB) de l'Union européenne, n'a pas remporté l'adhésion des États membres et n'a pas permis de surpasser les divergences maintenant bien connues entre ceux-ci. Si les conclusions quelque peu lapidaires du Conseil européen ne cèdent pas à l'inquiétude, le calendrier des négociations s'avère toutefois de plus en plus contraint pour permettre un démarrage des programmes opérationnels dès janvier 2021. En confiant désormais le suivi des négociations au président du Conseil européen, les États membres ont voulu opter pour un changement de méthode, dont nous espérons qu'il portera rapidement ses fruits. Un sommet dédié à ces négociations pourrait se tenir au début de l'année prochaine. Madame la secrétaire d'État, vous avez été interrogée à plusieurs reprises, y compris lors du dernier débat préalable au Conseil européen, sur les « lignes rouges » du Gouvernement en matière de calibrage du budget européen, qu'il s'agisse global ou des sous-enveloppes dédiées aux principales politiques communes. Or la France ne s'est pas encore engagée formellement sur le budget européen exprimé en pourcentage du RNB qu'elle souhaite défendre. Pourriez-vous, madame la secrétaire d'État, clarifier la position de la France quant au niveau minimal que devrait atteindre le budget européen pour les années 2021 à 2027 ? De plus, si les négociations semblent traîner depuis plusieurs mois, les données de l'équation ne cessent d'évoluer. Alors que les États membres ne parviennent à s'accorder ni sur le niveau global du budget ni sur les priorités à financer, la Commission européenne vient de présenter sa feuille de route pour un « pacte vert », incluant notamment un « mécanisme pour une transition juste » pouvant engendrer jusqu'à 100 milliards d'euros d'investissements. Madame la secrétaire d'État, comment la création de ce nouveau fonds s'articulera-t-elle avec les négociations budgétaires en cours ? financer de nouvelles dépenses, ce fonds ne vise-t-il pas à compenser les coupes budgétaires annoncées pour la politique de cohésion ? Un autre instrument budgétaire à financer a vu le jour depuis le début des négociations relatives au prochain cadre financier pluriannuel, il y a dix-huit mois. Il s'agit de l'instrument budgétaire de convergence et de compétitivité, auparavant désigné comme le « budget de la zone euro », dont le président de la commission des finances, Vincent Éblé, que je remplace ce soir, a dénoncé le manque d'ambition à plusieurs reprises. Si son financement devra être prévu par le cadre financier pluriannuel, les conclusions sommaires du sommet de la zone euro du 13 décembre témoignent de la difficulté à avancer collectivement sur ce dossier. Enfin, le Conseil européen a permis aux États membres de faire le point sur l'avancée du Brexit, juste après que les élections législatives britanniques ont confirmé le soutien de la majorité Il est vrai que les États membres ont accueilli avec un soulagement certain l'issue de ce scrutin, qui permet de clarifier la majorité à la Chambre des communes et de confirmer la tenue d'un Brexit d'ici à la fin Pour autant, un nouveau front de négociations s'ouvre désormais, et il n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit maintenant de déterminer nos relations futures avec le Royaume-Uni. Si le Conseil européen a réaffirmé son souhait d'établir des relations aussi étroites que possible avec le Royaume-Uni, le Gouvernement britannique a confirmé qu'il ne souhaitait pas une extension de la période de transition, imposant ainsi qu'un accord commercial soit trouvé d'ici à la Madame la secrétaire d'État, comment un accord commercial permettant de garantir des relations étroites et équitables peut-il être trouvé dans un temps aussi contraint ? Ne craignez-vous pas que seul un accord soit conclu, au risque de favoriser une forme de dumping social et fiscal outre-Manche ? Vous nous préciserez également les contours du mandat de négociation qui devrait être proposé par la Commission européenne. La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, lors du débat préalable au Conseil européen, nous nous étions concentrés sur les enjeux budgétaires. la négociation du cadre financier pluriannuel de l'Union figurait en bonne place dans l'ordre du jour de ce sommet. La présidence finlandaise avait d'ailleurs publié, début décembre, un nouveau cadre de négociation chiffré, auquel chacun des groupes politiques du Sénat avait pu réagir lors de ce débat préalable. Pourtant, le Conseil européen des 12 et 13 décembre ne s'est pas attardé sur ce sujet. La cacophonie entre les États membres, tant sur la question des ressources propres que sur la ventilation des dépenses, est apparue telle que le cadre financier pluriannuel fera finalement l'objet d'un sommet extraordinaire en C'est en fait l'ambition européenne pour le climat qui aura focalisé l'attention lors de ce Conseil européen et qui sera, de ce fait, au coeur de mon propos en introduction à ce débat. Il faut dire que la présidente de la Commission européenne avait habilement présenté la veille au Parlement européen les grandes lignes du Pacte vert qui doit permettre d'assurer la transition climatique et écologique de notre continent. Le Conseil européen a donc été conduit à prendre note de cette communication. Surtout, il a fixé à l'Union européenne l'objectif d'atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050, conformément aux objectifs déterminés par l'accord de Paris. de Paris. Même si cette décision résulte de longs mois de préparation pour convaincre les États membres de l'endosser, elle n'était pas facile à prendre. La Pologne, très dépendante du charbon, est restée récalcitrante, si bien que le Conseil européen indique, dans ses conclusions, qu'un État membre, à ce stade, ne peut s'engager sur cet objectif. L'Union évite ainsi d'être prise en otage par un seul État membre qui faisait monter les enchères pour prix de son ralliement.

alors même que la COP25 réunie à Madrid n'a pas tenu ses promesses. En effet, les parties à l'accord de Paris ont reporté à plus tard le traitement des questions qui fâchent. Nous pouvons aussi nous féliciter de la confirmation expresse par le Conseil européen du respect du principe de neutralité technologique pour parvenir à l'objectif de neutralité carbone. La liberté de chaque État de choisir son mix énergétique est donc préservée. Nos voisins tchèques, hongrois et slovaques ont même obtenu qu'à ce titre le nucléaire soit mentionné dans les conclusions du Conseil européen. En tant qu'élu de la Manche, je tiens à les saluer tout particulièrement. Je vois que je fais plaisir à mon collègue André Gattolin

C'est une avancée importante : pouvez-vous nous dire, madame la secrétaire d'État, si elle a des chances d'être consacrée dans le texte final, puisque le Parlement européen aura son mot à dire ? Chacun sait la sensibilité de ce dernier à ces questions. Enfin, je me réjouis que le Conseil européen se soit attaché à souligner la nécessité, pour l'Union, de veiller à ce que sa transition climatique n'entame pas sa compétitivité- au sein de cette assemblée, madame la secrétaire nous y sommes extrêmement attachés. C'est pourquoi il appuie le projet de mécanisme d'inclusion carbone aux frontières. Ce mécanisme, que vous nous aviez clairement présenté lors du débat préalable à ce Conseil européen, est vertueux. Tout en étant compatible avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), il doit permettre de corriger l'écart entre nos normes environnementales et celles des pays dont nous importons les biens. C'est donc une nouvelle politique commerciale très offensive qui se profile pour l'Union européenne

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, si le Brexit n'était pas à l'ordre du jour du Conseil européen, on peut néanmoins se réjouir de la clarification apportée par le résultat des élections britanniques à la Chambre des communes. La large victoire des conservateurs ouvre théoriquement la voie à une sortie négociée du Royaume-Uni le 31 janvier prochain. En attendant, nous savons déjà que ce départ va priver le budget européen de 12 milliards d'euros chaque année. J'en viens ainsi au prochain cadre financier pluriannuel, qui a une nouvelle fois occupé une partie des discussions du Conseil, en particulier la dernière proposition de la présidence finlandaise d'un budget s'établissant à 1 087 milliards d'euros pour les années 2021 à 2027.

Cette proposition suppose une baisse des moyens de l'ordre de 47 milliards d'euros sur sept ans. Peut-on s'en satisfaire, alors même qu'il est demandé à l'Union européenne de poursuivre ses politiques traditionnelles tout en assumant de nouvelles priorités, en particulier en matière de sécurité, de défense et de gestion des migrations ? ? Pour sortir de cette équation difficile, je crois qu'il faut dépasser le débat entre les moins-disants et les mieux-disants en matière de contributions nationales et se pencher sur les ressources propres, qui ont le mérite, je le rappelle, de ne pas peser sur le contribuable européen. Mon groupe est favorable à ce que ces ressources propres soient modernisées et accrues. Il le faudrait d'autant plus que, parmi celles-ci, le produit des droits de douane est de moins en moins dynamique avec la multiplication des accords de libre-échange. Pour alimenter le budget, l'idée de créer une taxe carbone aux frontières est pertinente ; je salue, madame la secrétaire d'État, votre détermination à la faire avancer. Outre que le mécanisme s'inscrirait dans la politique de l'Union pour la neutralité climatique, sa mise en oeuvre induirait un rapport d'équité entre nos entreprises européennes, soumises à des normes strictes, et celles celles des pays tiers qui ne sont pas contraintes par les mêmes exigences. Attendons cependant de voir ce que l'OMC pensera de tout cela. Je m'inquiète en revanche du manque de soutien de plusieurs États membres à la création d'une taxe sur les activités numériques, que la France souhaite ardemment.

En effet, en dehors du caractère de ressource propre que le produit de la taxe numérique pourrait avoir, selon la théorie Mundell-Fleming, une zone monétaire n'est optimale qu'à plusieurs conditions, dont un encadrement de la concurrence fiscale et sociale. Mais c'est là un autre débat de la ventilation des crédits, mes chers collègues, je ferai quelques observations sur la proposition finlandaise. Je note avec satisfaction l'effort de 10 milliards d'euros consenti au bénéfice de la politique agricole commune (PAC), même si son fléchage au profit du second pilier est discutable, compte tenu des attentes des agriculteurs en matière de soutiens directs. Par ailleurs, je m'interroge, comme plusieurs de mes collègues, sur la diminution de 6 milliards d'euros du budget du Fonds européen de la défense. Cette coupe est un mauvais signal au moment où l'on répète souvent que l'Europe doit garantir son autonomie stratégique et capacitaire. La semaine dernière encore, ici au Sénat, dans le cadre du débat que nous avons consacré à l'OTAN, le RDSE, à l'instar d'autres groupes, a rappelé son souhait de voir renforcer l'Europe de la défense. Le ministre des affaires étrangères a lui-même souligné la nécessité, pour les États membres, d'être plus proactifs et de prendre davantage leurs responsabilités pour assumer la sécurité collective. Je sais que le Gouvernement français déplore cette baisse. Nous comptons sur vous, madame la secrétaire d'État, pour la contester. Dans le prochain cadre financier pluriannuel, il faudra aussi tenir compte de l'enveloppe dédiée au budget de la zone euro, soit 14 milliards d'euros pour le nouvel instrument budgétaire de convergence et de compétitivité. À cet égard, le Président de la République aurait souhaité davantage. Si cela ne suffit pas, quel type de financement additionnel peut-on imaginer ? Cet instrument pourrait constituer un véritable pare-feu à un éventuel choc asymétrique. En cas de crise, les réponses budgétaires ne suffisent bien souvent qu'à panser les plaies. Il faut donc encourager les réponses macroéconomiques au sein de la zone euro. Dans le même esprit, il faut absolument débloquer le dossier du troisième pilier de l'union bancaire.

On ne peut que souscrire à cet horizon, car pour reprendre une formule de l'ancien ministre Hubert Védrine, il y a « la nécessité vitale de garder la terre habitable ». Est-il utile de rappeler que l'urgence s'ajoutera à l'urgence si l'on ne prend pas les bonnes décisions dès aujourd'hui ? Dans cette perspective, le Pacte vert pour l'Europe récemment dévoilé par la commissaire Ursula von der Leyen va dans le bon sens. Sans entrer dans le détail, je dirai simplement que si l'objectif de neutralité climatique doit être partagé par tous les États membres, le rythme pour l'atteindre l'atteindre doit être différencié afin de lever les inquiétudes de certains partenaires, au premier rang desquels la Pologne. À cet égard, la mention, dans les conclusions du Conseil européen, du droit de décider de son mix énergétique, apporte une flexibilité souhaitable. Pour le financement à long terme de cette politique, le fonds de transition juste de 100 milliards d'euros sera-t-il suffisant ? Nous attendons des clarifications de l'exécutif européen sur la répartition de ce financement. Mes chers collègues, le groupe RDSE, attentif à l'approfondissement du projet européen, observe avec intérêt les quelques décisions de ce Conseil européen qui permettront, je l'espère, d'améliorer la réponse collective aux grands défis qui nous attendent.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le Conseil européen qui s'est tenu la semaine dernière était le premier depuis le renouvellement des principales institutions de l'Union européenne. Pour Charles Michel, le nouveau président du Conseil européen, cette première réunion, essentiellement consacrée aux enjeux climatiques et au prochain cadre financier pluriannuel, ne sera à coup sûr pas la dernière, tant les points de désaccord entre États membres sont encore nombreux et délicats à arbitrer. On peut bien sûr se féliciter de ce que les dirigeants européens aient approuvé l'objectif de rendre l'Union européenne neutre pour le climat d'ici à 2050, même si la Pologne estime, à ce stade, qu'elle ne peut s'engager à mettre en oeuvre cet objectif. Le Pacte vert présenté par la nouvelle Commission, qui porte sur un investissement de 1 000 milliards d'euros, devrait être le principal levier de cet ambitieux projet qui ferait de l'Union européenne le seul grand acteur mondial à se conformer strictement aux accords de Paris sur le climat. Après la piètre COP25 qui se déroulait en parallèle à Madrid, il est bon que l'Union ait, lors de ce Conseil européen, affirmé ses ambitions climatiques et esquissé les moyens envisagés pour leur Mais, là encore, des objectifs proclamés à leur atteinte, la route risque d'être longue et parsemée d'embûches. La première d'entre elles concerne l'adoption du prochain cadre financier pluriannuel de l'Union. La Commission souhaite qu'à terme

Pour autant, même échelonnée sur plusieurs années, la mutation risque d'être rude et se heurtera à coup sûr à nombre de réticences, d'autant que le cadre financier présenté par la présidence finlandaise quelques jours avant la tenue du Conseil européen est très loin d'avoir fait l'unanimité. C'était bien évidemment prévisible. C'est en effet le sort attendu de tout « texte martyr » que de subir le martyre. Or la proposition finlandaise était bel et bien un texte martyr, et il eût été étonnant que ses arbitrages assez abrupts entre les différentes politiques politiques de l'Union obtinssent l'assentiment des États membres. En la matière, le président Charles Michel aura, il le sait, encore beaucoup à faire dans les mois à venir pour accorder les violons avant d'entendre retentir une triomphale au dernier étage du Berlaymont

Le premier message, c'est que le Conseil n'est pas prêt à procéder à une augmentation très substantielle du budget de l'Union. Avec 1 087 milliards d'euros proposés pour le cadre financier entend rester au même niveau budgétaire que l'Union à vingt-huit au cours du CFP précédent, soit bien en deçà des propositions de la Commission européenne, et plus encore de celles du Parlement européen. On peut le regretter, mais, en matière d'élargissement du budget européen, il en va, à notre sens, probablement de même qu'en matière d'élargissement tout court de l'Union : il convient de s'assurer du bon fonctionnement et de l'équité des procédures aujourd'hui à l'oeuvre avant de se lancer tête baissée dans l'aventure. Pour pallier le départ du Royaume-Uni, les pays contributeurs nets vont devoir mettre encore un peu plus la main à la poche, et cette solidarité budgétaire entre États membres doit s'accompagner d'une solidarité politique de la part des États bénéficiaires, en matière de respect tant des engagements pris dans les domaines de la lutte contre la corruption et de l'indépendance de la justice que des normes sociales et environnementales de l'Union. C'est là le deuxième message adressé par la présidence finlandaise en cette fin de mandat : celui de la conditionnalité de l'attribution de certains fonds européens, en particulier dans le domaine de la politique de cohésion, au respect effectif de certains principes fondamentaux de l'État de droit et de la lutte contre le détournement des aides allouées. allouées. Certains pays bénéficiaires nets, qui réclament une augmentation importante du budget européen, sont ici très directement visés. La solidarité des régions riches de l'Union envers celles qui le sont moins fait partie des principes fondamentaux de l'Union. Mais, il faut le dire très clairement, il ne s'agit en rien d'un droit de tirage automatique, sans exigence respect des engagements pris en contrepartie par les pays bénéficiaires. Il est bon de le rappeler, l'Union européenne n'a pas qu'un objet économique ; elle est également une communauté de valeurs et de pratiques entre des pays aux règles démocratiques qui s'engagent à respecter et à faire vivre l'État de droit.

enfin à entrer dans les moeurs des instances de l'Union ; c'est là une très bonne chose. Le troisième message fort du Conseil s'adresse à une partie des États les plus prospères de l'Union : il annonce sa volonté d'en finir avec constituent les « rabais sur le rabais », qui font que certains pays compensent moins qu'ils ne le devraient le fameux rabais accordé dans les années quatre-vingt au Royaume-Uni sur sa contribution nationale au budget de l'Union. Avec la mise en oeuvre du Brexit, entérinée par les élections du 12 décembre dernier, ce système complexe de compensation n'a plus de raison d'être. Parce que ces États devront mécaniquement contribuer davantage au budget de l'Union, cela les rend évidemment peu enclins à accepter de dépasser le niveau de 1,07 % du RNB proposé par la Finlande pour le prochain cadre financier pluriannuel. C'est là précisément que la question du futur cadre budgétaire européen croise celle de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui s'ouvrira au printemps prochain. Ce n'est pas seulement le financement effectif du Pacte vert qui est en cause ; c'est aussi celui des nouvelles politiques voulues par la nouvelle Commission, en matière tant de sécurité et de défense que de politique spatiale ou d'investissements dans les nouvelles technologies.

l'Union semble ne pas être en mesure d'augmenter substantiellement son budget, s'agit-il là, madame la secrétaire d'État, d'une alternative envisagée, qui consisterait à s'appuyer sur une action coordonnée de plusieurs États européens à travers leurs budgets et sur une politique de la concurrence moins dogmatique pour donner à notre continent les moyens de relever les défis du futur qui semblent désormais avoir été clairement identifiés par la nouvelle Commission ? La parole

d'un fonds pour la transition juste doté de 100 milliards d'euros, mais pour quoi faire exactement ? À quoi et à qui va servir cet argent ? Sur quels critères les fonds seront-ils accordés ? Pour quels projets ? Sous le contrôle de qui ? de qui ? S'il s'agit de financer les mêmes stratégies d'entreprise, le même modèle de développement économique et social au service des mêmes exigences de rentabilité

Il n'y a pas de transition juste sans nouveaux critères de financement. Le fonds de transition juste doit être géré de manière transparente. À cet égard, quel mécanisme précis de transparence le Gouvernement est-il prêt à mettre en place pour les projets qui seront financés en France avec cet argent ?

le Président de la République déclare vouloir tout à la fois renouer le dialogue avec la Russie et européaniser l'OTAN en faisant de la défense européenne son pilier européen, alors même que la déclaration finale du sommet de l'OTAN désigne la Russie comme la principale menace. Comment allons-nous régler cette contradiction ?

sont les mêmes qui signent une déclaration finale, au sommet de l'OTAN, avec la Turquie, alors que l'accord entre la Turquie et la Libye pose de très sérieux problèmes à deux États membres de l'Union européenne : la Grèce et Chypre.

ce Conseil européen, le dernier de 2019 et le premier des nouveaux visages européens, aura été marqué une nouvelle fois par le Royaume-Uni. La question du Brexit, ombre orageuse dans le ciel bruxellois depuis plusieurs mois, semble s'éclaircir, et 2020 pourrait bien être l'année du dénouement. Les Britanniques ont donné une large majorité à Boris Johnson, faisant le choix de rendre le Brexit réalité. Ainsi, le 1 février prochain, nous pourrions n'être que

Le risque d'un Brexit dur n'est pas écarté. Le Président de la République a été clair, évoquant le maintien d'une relation étroite, notamment en matière de commerce et de défense. Il a aussi rappelé que la protection et la garantie des intérêts européens sont une priorité.

Le Conseil a d'ailleurs chargé la Commission européenne de présenter un projet de mandat global. La nouvelle phase de négociations est cruciale pour nous tous. Madame la secrétaire d'État, les lignes rouges européennes, qui ont été tenues jusque-là, seront-elles respectées sous ce mandat ? ? Pouvez-vous nous assurer que la volonté de nouer une relation étroite avec le Royaume-Uni ne nous empêchera pas de garder notre unité et de protéger nos intérêts face à ce pays allié qui souhaite tout de même se désolidariser d'une construction inédite au regard de l'histoire ? Ce Conseil européen sera aussi à intégrer à l'échelle de l'histoire. La question du changement climatique a été mise à l'honneur. Nous ne pouvons que nous féliciter de l'obtention d'un accord sur l'objectif de la neutralité carbone de l'Union européenne en 2050, et ce dans la dernière semaine de la COP25 et de la présentation d'un ambitieux par la Commission européenne. Le calendrier proposé par cette dernière est exigeant

Je tiens aussi à saluer le fait que l'objectif de la neutralité carbone en 2050 prenne en compte les questions sociales, mais également celle de la compétitivité de l'Union européenne. À ce propos, le mécanisme d'ajustement des émissions de carbone aux frontières est intéressant. Quelle est la position de la France sur ce sujet cher au Gouvernement ? La question de la sécurité énergétique a aussi été abordée. Elle est essentielle. Nous croyons à un mix énergétique efficace et décarboné faisant toute leur place aux sources d'énergie renouvelables, ainsi qu'au nucléaire.

propre transition. Ne serait-il pas plus efficace d'orienter les aides octroyées à la Pologne dans une perspective de transition énergétique respectueuse des volets sociaux et économiques, plutôt que de casser notre politique du consensus et de créer un précédent ? De mémoire récente, les mécanismes d'et les précédents n'ont pas vraiment prouvé leur efficacité au sein de l'Union européenne. Enfin, viser la neutralité carbone suppose un budget. Or de budget, il a été peu question lors du sommet européen. Bien sûr, il y a eu des déclarations concernant la nécessité d'un budget solide pour assurer une transition efficace et équilibrée. Nous avons entendu affirmer une nouvelle fois que 25 % du prochain cadre financier pluriannuel devrait être consacré à la lutte climatique, mais les discussions ont été remises à plus tard ... Nous l'avions noté avant le Conseil européen, le cadre de négociation du cadre financier pluriannuel proposé par la présidence finlandaise est loin de faire l'unanimité.

ce qu'il en est des négociations sur le budget de la PAC ? Vos objectifs concernant le premier pilier seront-ils tenus ? Enfin, je souhaite saluer les discussions au sujet de la tenue d'une conférence sur l'avenir de l'Europe. L'après-Brexit et le début de la nouvelle mandature européenne sont propices à une grande réflexion sur notre système et sur notre avenir. Je forme le souhait qu'une consultation citoyenne soit engagée durant le processus. Une partie de l'avenir de l'Europe se jouera en 2020 sur les questions du budget et de la transition, ainsi

madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le Conseil européen qui vient de se conclure était stratégique à plusieurs égards. Il parachève une année marquée par les incertitudes du Brexit, des élections européennes déstabilisant le institutionnel et par de fortes attentes quant à l'action de l'Union européenne. À ce titre, la France a joué un rôle moteur, illustrant bien une citation de Victor Hugo toujours d'actualité L'Europe ne peut être tranquille tant que la France n'est pas contente. » En effet, cette année, sur de nombreux sujets, la France s'est distinguée par un positionnement singulier, qu'il s'agisse de défendre une souveraineté européenne à construire, de repenser une politique commune de concurrence obsolète ou bien d'interroger une stratégie d'élargissement qui ne peut pas constituer la seule perspective pour le voisinage de l'Union. Ce Conseil européen n'a pas fait exception à cet égard, et nous pouvons nous en féliciter. J'aimerais tout d'abord insister sur l'importance de ce sommet. Avec une nouvelle équipe et l'esquisse de nouveaux projets ambitieux à court, moyen et long termes, l'Europe revient à un agenda positif, alors que celui de la précédente Commission avait été davantage dicté par les nombreuses crises qu'elle avait dû assumer. Au coeur de ce nouvel agenda réside l'objectif de faire de l'Union européenne le premier continent neutre en matière d'émissions Je salue une telle ambition, reflétant un pouvoir d'initiative retrouvé, qui permettra à l'Europe- j'en suis sûr -d'orienter les grandes transformations que connaît notre monde. Relever ce défi nécessitera des efforts communs, consentis au travers d'une solidarité accrue. Ce sera une occasion idéale de réaliser un travail d'introspection. D'une part, la solidarité sera essentielle au regard de la diversité des mix énergétiques, sachant que l'Union s'effectuera nécessairement dans la diversité. À ce titre, la défense de la transition écologique ne doit pas se réduire à des mesures punitives envers nos voisins de l'Est. Il s'agit de considérer l'effort de transition comme offrant de vraies perspectives, qui doivent être socialement justes, démocratiquement acceptables et territorialement différenciées. D'autre part, les objectifs du imposent de « mettre en place un cadre facilitateur » comprenant « un soutien et des investissements adaptés À cet égard, je suis convaincu que faciliter les investissements dits « verts » doit se faire en permettant aux États membres de les extraire du pacte de stabilité et de croissance, comme l'a suggéré notamment le nouveau commissaire à l'économie, Paolo Gentiloni.

dernier. Je tiens à saluer la prise en compte d'un critère climatique dans les accords commerciaux et la décision de l'Europe de ne plus contracter d'accords commerciaux avec des puissances qui ne sont pas signataires de l'accord de Paris. de l'accord de Paris. L'agenda positif que j'évoquais précédemment permet de comprendre les tensions et les enjeux entourant le prochain cadre financier pluriannuel. Bruxelles, comme il est coutume de l'appeler, ne saurait faire plus avec moins. Les discussions portent à l'heure actuelle tant sur le niveau du budget que sur les arbitrages entre les politiques dites « historiques » et les politiques nouvelles, en matière climatique, numérique et de défense. si le Conseil européen n'a pas été l'occasion d'obtenir des avancées sur le sujet, permettez-moi de vous alerter sur les risques de ce futur budget. En effet, s'il est indéniable que le soutien à l'innovation et aux politiques numériques est indispensable, conjugué à la diminution des fonds destinés à l'agriculture et à la pêche, serait potentiellement susceptible de venir creuser les disparités régionales, alors même que l'on constate un écart économique de plus en plus important entre les capitales et les périphéries, en dépit des tentatives de réajustement. de réajustement. Une nouvelle dynamique est insufflée à l'Europe. Nous ne pouvons que nous en réjouir. L'Europe ne souhaite plus se contenter de réagir aux crises ; elle veut dorénavant tracer sa propre trajectoire. Cela démontre que son histoire est celle d'un destin voulu. la suite des élections européennes du mois de mai dernier, certains voient un Parlement divisé et fragmenté. Pour ma part, j'y vois un Parlement qui a démontré qu'il entendait, lui aussi, assumer un rôle actif et ne pas se contenter de celui de chambre d'enregistrement. Le Parlement européen restant la seule institution européenne directement élue par les citoyens, j'accueille une telle position avec bienveillance. le constat d'une bataille institutionnelle, et alors que la nouvelle Commission européenne a pris ses fonctions avec un mois de retard, le Conseil souhaite repenser le processus des nominations à l'échelon européen. Il propose à ce titre d'organiser dès le mois de février 2020 une réflexion sur le fonctionnement des institutions : c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe.

Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous éclairer sur les enjeux de cette conférence, sur les ambitions du Gouvernement à cet égard et sur le rôle qui sera accordé aux parlementaires nationaux nationaux ? En raison de leur ancrage et de leur présence sur nos territoires, ceux-ci restent des relais indispensables pour vulgariser une telle conférence et inciter nos concitoyens à y participer pleinement.

Enfin, alors que l'Union a donné son feu vert à l'« Airbus des batteries », en autorisant sept États à subventionner à hauteur de 3,2 milliards d'euros le consortium de dix-sept entreprises créé pour l'occasion, quelles sont les ambitions du Gouvernement en matière de politique européenne de concurrence après le rejet regrettable, en février dernier, de la fusion entre le français Alstom et l'allemand Siemens ? La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le Conseil européen qui s'est tenu la semaine dernière était un rendez-vous important.

réunion importante marque en outre le coup d'envoi du nouveau cycle institutionnel ouvert avec les élections européennes et la mise en place de la Commission von der Leyen. Avant la tenue de ce sommet, la présidence finlandaise avait formulé le voeu que la nouvelle donne fasse « souffler un vent de fraîcheur » sur le Conseil, lui permettant ainsi de surmonter ses divergences, sur le plan tant climatique que budgétaire. Mais l'événement le plus significatif du 12 décembre se déroulait davantage au Royaume-Uni qu'à Bruxelles. En effet, sauf énième rebondissement, la large victoire électorale des conservateurs ouvre enfin la voie à l'adoption de l'accord de retrait. Il ne s'agit en aucune manière d'un point final apporté au Brexit, eu égard à la nécessité de retisser les liens rompus avec le Royaume-Uni et de préserver autant que possible une relation stratégique, commerciale, sécuritaire et géopolitique vitale tant pour les Britanniques que pour les Européens. C'est finalement sur cet enjeu que portera la véritable négociation du Brexit, et ne nous y trompons pas : elle sera aussi exigeante que longue, certainement beaucoup plus longue que la période de transition définie par l'accord de retrait. Nous sommes donc loin d'en avoir fini avec le Brexit. Durant la nouvelle phase qui va s'ouvrir, les Européens devront veiller à demeurer aussi unis qu'ils l'ont été jusqu'à maintenant sous la conduite de Michel Barnier.

et « invite son président à faire avancer les négociations en vue de parvenir à un accord final ». Voilà tout ce qui ressort des discussions. Cela illustre à quel point les positions des uns et des autres restent figées. Comme on pouvait le supposer, la boîte de négociation chiffrée proposée par la présidence finlandaise, en baisse de 50 milliards d'euros par rapport à la proposition de la Commission, n'a pas permis de rapprocher les points de vue. Les divers groupes d'États membres qui se sont constitués, et qui parfois s'entrecroisent, autour des grands enjeux de ce CFP ne semblent pas encore décidés à bouger. Dans ces conditions, on peut craindre que l'issue de la négociation ne permette pas à l'Union de disposer, à partir de 2021, d'un budget réellement à la hauteur de tous les objectifs. Deux points me paraissent particulièrement inquiétants : d'une part, le niveau toujours insuffisant, malgré la revalorisation proposée pour le deuxième pilier, du budget de la PAC ; d'autre part, la baisse drastique envisagée de la dotation pour le Fonds européen de la défense. Madame la secrétaire d'État, malgré une ambition vraisemblablement bridée, sur ces deux sujets, par une enveloppe globale contrainte, pensez-vous, au vu de vos discussions avec vos homologues,

Les conclusions du Conseil sont un peu plus loquaces concernant la question climatique. Néanmoins, la situation n'est pas si différente de celle du mois de juin, quand l'objectif de la neutralité carbone d'ici à 2050 n'avait pas pu être endossé en raison de l'opposition de quatre États membres particulièrement dépendants du charbon. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un : la Pologne. Il est toutefois raisonnable d'espérer que des discussions plus approfondies sur le présenté la semaine dernière, mais aussi sur le CFP, s'agissant notamment du fonds pour une transition juste, seront de nature à convaincre Varsovie de se joindre au reste de l'Union Notre continent s'apprête donc à passer à la vitesse supérieure en matière climatique et à accélérer sa transition écologique. Après la définition des objectifs globaux, il convient désormais d'établir la stratégie.

ont de fortes incidences sur l'environnement physique, mais également sur le monde vivant et sur l'activité économique dans nos massifs. Mais, en montagne comme ailleurs, si la transition écologique exige des efforts colossaux pour transformer en profondeur notre économie et l'ensemble de nos activités, elle doit constituer un véritable levier de développement. Dans le cas contraire,

Elle réussira si nous sommes en mesure d'en faire aussi un levier de création d'emplois et de valeur ajoutée. Toute politique climatique ambitieuse devra donc nécessairement aller de pair avec une politique industrielle intelligente et ambitieuse qui prenne pleinement en compte toutes les réalités de l'économie du XXI siècle. siècle. Je le souligne une nouvelle fois, dans le cadre de la grande transformation de nos politiques publiques, nous aurons un impérieux besoin de conditions de concurrence équitables à l'échelle mondiale pour préserver notre compétitivité. Faire de l'Europe une île décarbonée au milieu d'un monde qui, lui, n'évoluerait pas ne serait cohérent ni économiquement ni écologiquement. L'introduction d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Europe qui rééquilibrerait les conditions de l'échange international et découragerait les fuites de carbone, notamment des délocalisations vers les pays moins exigeants en matière climatique,

Pour relever cet immense défi, gardons à l'esprit que si l'ambition est non plus une option, mais une nécessité, elle ne pourra se concrétiser qu'en combinant deux qualités aussi fondamentales que complémentaires des Européens : la créativité et le pragmatisme. Très bien

Il n'y a pas d'économie durable sans finances durables. Ces éléments, qui devront être progressivement améliorés, sont essentiels. Il faudra aussi que l'Union européenne pèse pour que les critères de Bâle III évoluent afin de tendre vers un « Bâle vert

je veux saluer le travail de la présidence finlandaise pour satisfaire aux exigences du traité de Lisbonne s'agissant de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme.

le Conseil européen de la semaine dernière avait un ordre du jour chargé, avec en toile de fond les élections législatives britanniques. La victoire très nette de Boris Johnson met fin à l'incertitude qui régnait quant à une mise en oeuvre effective du Brexit. Sauf énorme surprise, le Royaume-Uni quittera bel et bien l'Union européenne d'ici au 31 janvier prochain. Le Premier ministre Johnson a désormais une majorité très confortable, et surtout un mandat clair pour négocier à Bruxelles, ce qui rééquilibre le rapport de force entre le Royaume-Uni et l'Union Il importe donc que les vingt-sept restent unis dans les prochains mois, comme ils l'ont toujours été depuis le résultat du référendum britannique. C'est en effet une nouvelle phase délicate qui va s'ouvrir le 1 février 2020, date à laquelle les Vingt-Sept entameront la négociation de leur futur partenariat stratégique avec Londres. Cette nouvelle relation devra bien entendu être la plus étroite possible. Mais elle devra aussi, et surtout, être fondée sur un équilibre de droits et d'obligations, notamment pour éviter toute concurrence déloyale. Le mandat de négociation que la Commission européenne est en train de préparer devra être clair sur ce point Je me réjouis par ailleurs que Michel Barnier ait été nommé chef des futures négociations. Je fais confiance à son expérience et à ses talents de négociateur pour aboutir à un résultat juste et équitable. Le cadre financier pluriannuel pour 2021-2027 Les dirigeants de l'Union européenne ont invité le président du Conseil européen, Charles Michel, à faire avancer les négociations pour trouver un accord final. Toutefois, au regard des divergences profondes qui persistent, il ne sera sans doute pas évident de conclure en 2020 cette négociation, l'unanimité

pour sa capacité à assurer un niveau de vie correct à ses agriculteurs, pour sa souveraineté alimentaire et pour sa transition climatique. Il faut ensuite supprimer les rabais. Si cette suppression n'intervient pas à l'occasion du départ des Britanniques, elle ne se fera jamais revoir les ressources propres, en les mettant en rapport avec les objectifs ambitieux et nombreux que nos concitoyens assignent à l'Union européenne. Il faut enfin soumettre conditionner l'octroi des fonds européens, afin d'en faire des leviers utiles, au service notamment de l'État de droit. Le Conseil européen a aussi été marqué par des désaccords sur la future capacité budgétaire de la zone euro telle qu'elle a été élaborée par l'Eurogroupe. Le Portugal, en particulier, a ainsi manifesté son mécontentement au regard des coupes à venir dans le budget de la politique de cohésion post-2020. Le budget de la zone euro voulu par le Président de la République a décidément du plomb dans l'aile ! Le faible montant de ce budget- 17 milliards d'euros sur sept ans -ne révolutionnera pas l'économie européenne. J'ajoute que les pays du Nord s'opposent à la volonté française d'élaborer un accord intergouvernemental visant à mobiliser davantage de moyens nationaux pour accroître ce budget de l'eurozone. Bien sûr, nous partageons tous l'objectif de renforcer la résilience de la zone euro et la convergence économique en son sein. Pour l'atteindre, la durabilité des finances publiques, qui partout ailleurs en Europe se rétablit, doit demeurer une priorité. Au vu de son incapacité à redresser ses comptes publics et à transformer son économie, la France n'est sans doute pas l'avocat le plus indiqué pour défendre une telle évolution de la zone euro D'autres réformes semblent plus urgentes, comme l'achèvement de l'union bancaire et de l'union des marchés de capitaux. Cela permettrait de mieux absorber les chocs économiques en diversifiant les risques, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un budget commun de stabilisation. Sur ces dossiers, l'Union européenne Début décembre, les ministres de la zone euro n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur la mise en place du système européen de garantie des dépôts bancaires. Ces évolutions sont pourtant la base indispensable pour donner à l'euro sa vraie dimension dans les échanges internationaux. Dans le contexte géopolitique actuel, la monnaie unique doit être un instrument stratégique, capable de concurrencer enfin le dollar, grâce auquel les États-Unis exercent leur tutelle sur l'économie mondiale et sur leurs concurrents, l'extraterritorialité de leur droit. Je voudrais maintenant évoquer le projet de conférence sur l'avenir de l'Europe, voulu par le Conseil européen. Cette conférence devrait débuter en 2020 pour s'achever en 2022.

Si l'on ne peut qu'être d'accord avec le principe d'une telle concertation, je mettrai l'accent sur deux points de vigilance. D'abord, il ne faut pas oublier les territoires. Pour l'instant, l'échelon local semble absent des discussions. Or cette conférence doit être l'occasion, pour les institutions européennes, de marquer leur volonté de travailler avec les élus de terrain. Les exclure relèverait d'une vision de l'Europe dépassée, à l'heure où nos concitoyens ne se sont jamais sentis aussi éloignés du projet européen. Ensuite, il est prévu que la conférence aborde la question de la démocratisation des élections européennes, au travers notamment de la mise en place de listes transnationales par les familles politiques européennes. de faire des listes « hors sol » est un non-sens démocratique. L'affirmation du rôle du Parlement européen dans la fabrication des lois renforce le besoin d'un contrôle démocratique et d'une proximité avec les électeurs. L'élu doit leur rendre des comptes, mais encore encore faut-il qu'ils le connaissent ! C'est d'ailleurs ce manque de proximité qui explique l'importance du vote contestataire alors des élections européennes. N'en rajoutons pas ! Pour conclure, mes chers collègues, je ne voudrais pas oublier nos sapeurs-pompiers, avec qui l'on échange beaucoup sur le terrain en cette période de la Sainte-Barbe. Leur inquiétude est toujours vive concernant la directive Temps de travail, qui menace le statut de pompier volontaire. La France doit agir au niveau européen pour préserver le modèle de sécurité civile français. Exploiter les dérogations offertes par la directive de 2003, comme l'envisage le Gouvernement, ne suffira pas.

ouverte. Si nous trouvons, par exemple, un accord sur une taxe sur les transactions financières d'ici à 2022 ou à 2023, il faudra que l'on puisse brancher cette ressource sur le budget de la zone euro sans avoir à attendre 2027.

Bizet, Charles Michel a la volonté d'instaurer de nouvelles méthodes de travail. Nous avons déjà pu échanger sur ce sujet. Obtenir un consensus

de la production électrique en Europe ; le Parlement considère néanmoins que, en raison des déchets qu'elle génère, cette énergie nécessite une stratégie à moyen et long termes qui tienne compte des avancées technologiques- laser, fusion, etc. -visant à améliorer la durabilité du secteur. L'adoption de cet amendement peut, me

l'on commence à élaborer une directive sur l'engagement citoyen. Un certain nombre d'États membres sont très attentifs